La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Un laboratoire pharmaceutique américain et son partenaire allemand ont annoncé lundi de premiers résultats très encourageants concernant les tests de leur vaccin contre la covid-19. Cette nouvelle est incontestablement une lueur d'espoir dans le quotidien très assombri où sont plongés nos concitoyens depuis le début de l'année. Néanmoins, il faut rester prudent et rappeler que ces résultats sont des résultats intermédiaires ; un long processus est encore nécessaire avant une possible mise sur le marché. Cette attente, monsieur le Premier ministre, doit être synonyme d'anticipation. Le conseil scientifique a publié, le 9 juillet dernier, une note stratégique sur la vaccination contre la covid-19. C'est précisément sur cette stratégie que je souhaite vous interroger. Outre les défis de l'achat et de la production, nous en aurons plusieurs autres à relever, en matière de stockage et de distribution des doses, de mobilisation des personnels chargés de les administrer, mais aussi de définition des publics cibles. clair en effet que, malgré les injonctions de certains, toute la population ne pourra pas être vaccinée tout de suite. J'en viens par là même à une autre problématique : toute la population ne voudra pas être vaccinée. Les résistances sont importantes et les théories complotistes vont déjà bon train. Sans pédagogie, sans transparence, sans confiance, aucun vaccin ne viendra à bout de ce virus. J'aimerais donc savoir quelle est, à ce stade, la stratégie vaccinale du Gouvernement. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles.

de l'évaluation et du test de ce vaccin. Un certain nombre de tests doivent encore être effectués dans les semaines et les mois à venir, notamment pour évaluer les effets secondaires éventuels du vaccin. Viendra ensuite

puis de sa distribution au sein de la population. Vous avez dû noter que l'Union européenne a d'ores et déjà précommandé 200 millions de doses de ce vaccin auprès du laboratoire Pfizer.

Monsieur le ministre, en août dernier, vous affirmiez : « Nous sommes préparés à tout. » Depuis, tout le monde a pu constater que vous êtes plus dans l'improvisation que dans l'anticipation. Face à la deuxième vague, trois jours avant la rentrée de novembre, vous avez proposé un nouveau protocole sanitaire dit « renforcé ». Ce protocole s'est avéré inapplicable, voire inefficace, dans de nombreux établissements ; des lycéens et lycéennes se sont mobilisés et, après leur avoir répondu par la matraque, vous êtes tout de même convenu d'un ajustement substantiel en généralisant les demi-groupes dans les lycées. Mardi, le corps enseignant du secondaire s'est mobilisé pour demander un soutien renforcé de l'État, notamment dans les collèges. Du point de vue de la sécurité des enseignants, en effet, comment expliquer que l'obligation d'enseignement présentiel soit fixée à 50 % dans les lycées et maintenue à 100 % dans les collèges ?

au fondement même de notre contrat social, est fortement touché. Monsieur le ministre, les écologistes s'accordent avec la volonté de votre ministère d'assurer la continuité pédagogique, y compris dans la filière professionnelle ; la fermeture totale des établissements serait catastrophique. Mais votre gestion politique laisse encore trop d'enseignants, de personnels et d'élèves exposés à la pandémie. Ce que les enseignants et le personnel pédagogique appellent de leurs voeux, ce sont des mesures sanitaires spécifiques, mais surtout un soutien constant, notamment budgétaire, pour assurer pleinement leurs missions de service public dans un contexte certes complexe, mais appelé à durer. Les solutions existent ; elles sont mises en oeuvre dans d'autres pays recrutement massif de personnels enseignants, allégement des classes, investissement dans l'aération, soutien matériel au téléenseignement et, surtout, généralisation au collège des classes en demi-groupes. Monsieur le ministre, ma question est la suivante : allez-vous enfin rapidement mettre en oeuvre des mesures pour assurer la sécurité de tous les enseignants, personnels et élèves ?

est assez facile, pour une opposition, de souligner. Néanmoins, sur le terrain, nous avons réussi à ce que la plupart des écoles, des collèges et des lycées puissent continuer à fonctionner de façon aussi normale que possible.

Des mesures fortes ont été prises ; les établissements scolaires, lycées, collèges, écoles, restent ouverts pour assurer la continuité des enseignements et permettre aux élèves de préparer leur avenir malgré l'épidémie. Nous considérons que cette continuité éducative est essentielle, pour la raison évidente que je viens d'évoquer, mais aussi pour permettre aux parents de continuer à travailler, que ce soit à distance ou, dans les situations qui l'exigent, en présentiel. Pour autant, le risque sanitaire ne peut être éludé. Les établissements scolaires restent parmi les principaux lieux de diffusion du virus, en particulier lors des temps de restauration, durant lesquels les élèves de différentes classes sont en contact rapproché sans masques.

En effet, les études scientifiques sont formelles : si les adolescents sont moins menacés par la covid-19, ils sont susceptibles de transmettre le virus tout autant que les adultes, mais seraient asymptomatiques dans 50 % des cas. Ces informations nous conduisent à envisager des campagnes de dépistage massif parmi les lycéens et collégiens. Monsieur le ministre, vous avez annoncé le déploiement de un million de tests destinés aux enseignants. Pour que cette deuxième vague s'estompe rapidement, pour que les commerces de proximité et la vie sociale retrouvent leurs droits, pour que les effets du confinement ne soient pas neutralisés par la diffusion du virus dans les établissements scolaires et, par ce biais, dans les familles, nous pensons qu'il faut aller plus loin. La présidente de la région Île-de-France a d'ores et déjà annoncé la mise à disposition prochaine de 100 000 tests rapides dans les lycées afin de tester les personnels, ainsi que les élèves disposant d'une autorisation parentale. Le Gouvernement est-il prêt, monsieur le ministre, à envisager une campagne de dépistage généralisé auprès des lycéens et des collégiens, en partenariat avec les hôpitaux et les collectivités locales volontaires ?

Il est important que nous continuions à travailler avec les collectivités locales ; il est important aussi que chacun, dans son champ de compétences, fasse ce qu'il a à faire en matière de sécurité sanitaire. Rappelons que tout ce qui a trait au nettoyage, à l'hygiène, au brassage d'air, relève des collectivités locales, en étroite collaboration avec l'éducation nationale. J'appelle surtout les régions et les départements à être très actifs sur ces enjeux, y compris sur l'équipement informatique, domaine dans lequel nous avons fait de très belles avancées ces derniers mois et ces dernières semaines grâce à cette coopération. Concernant les tests, tout doit être fait, évidemment, en lien avec les agences régionales de santé. Les bonnes volontés sont bienvenues, mais nous avons les moyens de développer les tests nécessaires tout au long des prochaines semaines. Je suis confiant dans cet aspect des choses, et je rappellerai- cela a souvent été dit -qu'il n'y a pas une seule réponse

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Monsieur le ministre, le secteur de l'horticulture représente 3 300 entreprises et 20 000 emplois. Il pèse 1,64 milliard d'euros de chiffres d'affaires, mais l'horticulture française est aujourd'hui en danger de mort. En effet, le gouvernement français est le seul en Europe à avoir interdit la vente de fleurs coupées, tous créneaux de distribution confondus. Non contents d'avoir fermé nos fleuristes et commerces de proximité, vous interdisez aux grandes surfaces de vendre des fleurs, bien que celles-ci soient des produits agricoles. Dans mon département, l'entreprise Bigot, premier producteur de fleurs coupées en France, se bat au quotidien pour sa survie et celle de ses 200 emplois. Le recours au chômage partiel est faible, car il faut continuer à entretenir les cultures. Déjà fragilisée par le premier confinement, l'entreprise est très préoccupée par la gravité de la situation. Entendez-vous, monsieur le ministre, le cri de détresse de ces chefs d'entreprise et de leurs salariés ? Sans débouchés, l'entreprise Bigot détruit un million de tiges de fleurs par semaine. Pensez-vous que cela soit tenable, économiquement et humainement ? Le ministre de l'agriculture annonçait, en juin, un dispositif d'aide exceptionnelle de 25 millions d'euros pour le maintien de la filière. Aujourd'hui, pas un euro n'a été versé et ce dispositif ciblé n'est pas reconduit à l'occasion du second confinement, qui va causer des pertes abyssales. Sans intervention rapide, c'est la mort assurée pour les entreprises de ce secteur ! Monsieur le ministre, envisagez-vous de lever sans délai cette interdiction afin de sauver cette filière agricole ?

l'avez dit, les producteurs de fleurs coupées représentent environ 3 000 entreprises et plus de 20 000 salariés. Bien que leur activité n'ait jamais cessé pendant le confinement, ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation très difficile- nous le savons -, car ils continuent à produire et n'ont presque plus de débouchés de vente.

Notre objectif est de trouver des solutions pour que les producteurs puissent reprendre une activité de vente. Je me suis d'ailleurs entretenu à ce sujet mardi dernier avec Christiane Lambert, la présidente de la Mon collègue Julien Denormandie est à l'écoute de la filière pour lui apporter un accompagnement et une aide spécifiques, à l'exemple de ce qui a été fait avec les producteurs de pommes de terre, les producteurs de cidre et les brasseurs.

J'entends bien, monsieur le ministre, mais la fleur-tige est le seul produit agricole périssable qui aujourd'hui n'est pas autorisé à la vente. Ce qui n'est pas vendu va à la poubelle ! La fleur coupée doit rapidement réintégrer les circuits de distribution, à sa place habituelle, chez les fleuristes et au milieu des rayons de fruits et légumes, faute de légumes, faute de quoi nous allons tout droit vers un désastre économique pour tous ces producteurs qui oeuvrent au coeur de nos territoires et qui perpétuent une filière d'excellence. En campant sur vos positions, vous aurez la lourde responsabilité d'envoyer les salariés à l'abattoir et les entreprises à l'équarrissage

Depuis, peu de changements. Le recours aux ordonnances bat des records- c'est l'évitement permanent. Pour ce qui concerne l'état d'urgence sanitaire, le Sénat avait demandé que le Parlement puisse au moins approuver le recours au confinement- nouvelle fin de non-recevoir. Le transfert discret à Madagascar d'une couronne jusqu'à présent conservée au musée de l'Armée illustre une nouvelle fois ce mépris. En effet, le principe d'inaliénabilité des biens publics impose l'intervention du législateur pour tout transfert de ce type. Or nous avons appris le retour de cette couronne le lendemain de l'adoption par le Sénat du projet de loi entérinant le retour de certains biens culturels au Bénin et au Sénégal. Le prince dispose, le Parlement entérine ! Comment voulez-vous que le Parlement ne s'inquiète pas ? Des décisions cruciales ont été prises ce matin en conseil de défense,

Monsieur le Premier ministre, tout cela nous conduit malheureusement à devoir de nouveau vous poser la question que nous vous posions à votre entrée en fonctions : dans votre pratique institutionnelle, quand allez-vous permettre aux assemblées de jouer leur rôle ? Quand allez-vous

je me suis toujours employée à les respecter. Le travail que nous avons fait ensemble sur la restitution de biens culturels au Sénégal et au Bénin a été particulièrement fructueux ; je vous remercie d'ailleurs pour le vote unanime qui a été exprimé dans les deux chambres, grâce à un travail de concertation extrêmement fourni et approfondi. Pour ce qui concerne cet ornement de dais,

appelé les Malgaches à la révolte contre les colonisateurs français puis a reconnu sa défaite. Cet objet a donc surtout une valeur symbolique pour le peuple malagasy. Il ne s'agit en aucun cas d'une restitution,

fois expliquée en défendant le projet de loi de finances. Bien entendu, le principe d'inaliénabilité sera respecté. Si nous devions décider d'une restitution au gouvernement de Madagascar,

Comme cela a été dit il y a un instant, la découverte d'un vaccin contre la covid-19 fait naître une lueur d'espoir dans le climat pesant que nous continuons de traverser. Il est sûrement trop tôt pour confirmer tous les effets bénéfiques qui en sont attendus, mais la course est lancée ; il faut qu'à l'arrivée il y ait assez de doses pour tout le monde, avec une méthode et une approche permettant d'établir un climat de confiance ne laissant personne sur le bord de la route. Quelle que soit la manière dont s'organisera la diffusion du vaccin, il faut anticiper en tirant tous les enseignements des erreurs du passé. La Haute Autorité de santé a formulé, en juillet, ses recommandations pour la mise en place d'une stratégie vaccinale. Il faut donc maintenant se préparer. Et quand on voit les errements qui ont caractérisé la gestion du vaccin contre la grippe, je dois dire que nous ne sommes pas complètement rassurés Ma question est simple : puisqu'il faut anticiper l'arrivée sur le marché d'un vaccin contre la covid-19, que pensez-vous de notre proposition visant à mettre en place un pôle public de distribution du vaccin ? Et, en tout cas, quelles sont les dispositions que vous envisagez pour garantir la sécurité, la transparence, l'absence de spéculation des marchés financiers et, surtout, la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale du coût des doses de ce vaccin ?

recommandations pour l'élaboration d'une stratégie quant à la diffusion de ce vaccin. Elle aura de nouveau l'occasion de se prononcer et de formuler des recommandations qui nous permettront de définir la politique publique en la matière en tenant compte notamment de la disponibilité des vaccins. nous parlons du vaccin développé par un laboratoire en particulier, vous n'êtes pas sans savoir que d'autres laboratoires en sont à une phase avancée, autrement dit à la phase 3, du développement d'un vaccin- je pense à AstraZeneca, avec lequel la Commission européenne avait passé

deux doses pour Pfizer, une seule dose pour un certain nombre d'autres vaccins. Vous voyez qu'il y a encore un certain nombre de paramètres que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, et sur lesquels la Haute Autorité de santé aura à se prononcer afin d'élaborer cette stratégie que, comme nous, vous appelez de vos voeux. Le Gouvernement- je vous l'ai déjà dit

de conservation ; nous attendons les résultats des recherches. Permettez-moi enfin, monsieur le sénateur, d'ouvrir un petit peu le champ de votre question à l'international. La question de la disponibilité et de l'universalité

une embarcation de fortune transportant une vingtaine de passagers clandestins a chaviré au large de Cayenne. Si certains d'entre eux ont pu regagner le rivage par leurs propres moyens avant de disparaître dans la nature, il a fallu l'intervention de l'armée, de la Marine nationale et des pompiers pour porter secours aux autres occupants de l'embarcation, parfois très jeunes. Je tiens d'abord à saluer l'intervention rapide des militaires et des pompiers, qui ont permis d'éviter un véritable drame ; mais pour combien de temps encore ? Personne ne peut ignorer que la Guyane est victime d'une forte immigration, en raison de ses 378 kilomètres de littoral et de ses frontières fluviales avec le Suriname et le Brésil. À l'instar de ceux qui tentent de traverser la Méditerranée, beaucoup de clandestins entrent en Guyane au péril de leur vie. Nous avons déjà connu des drames. Bien qu'attachés à notre tradition d'accueil, nous ne pouvons plus absorber cet afflux massif. En effet, les structures d'accueil, comme les écoles, déjà en nombre insuffisant pour nos compatriotes, ne peuvent plus faire face. Les squats et bidonvilles, dans lesquels cohabitent l'insalubrité, la violence et souvent la mort, ne peuvent être le quotidien de nos compatriotes exaspérés. Monsieur le ministre, nous avons bien compris que les différentes mesures prises jusqu'à présent pour juguler l'immigration en Guyane n'ont pu pleinement porter leurs fruits et que les moyens mis en oeuvre pour garantir l'éloignement des personnes expulsées sont d'une portée limitée face à l'étendue de ces flux. C'est pourquoi je souhaiterais savoir, monsieur le ministre, comment le Gouvernement entend réaffirmer les pouvoirs régaliens de l'État en Guyane et ainsi mieux y contrôler l'immigration clandestine. Je vous remercie.

et Républicain. Nous venons d'apprendre la fermeture du site Bridgestone de Béthune. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer, au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, notre soutien et notre solidarité envers les 863 salariés qui vont être durement frappés par cette mesure. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le ministre, comme les petits commerçants ou les libraires, les personnels éducatifs, en plus de devoir faire face à la menace terroriste, payent eux aussi le manque de cohérence et l'impréparation du Gouvernement dans sa réponse à cette seconde vague. Il était indispensable d'assurer la continuité pédagogique durant le confinement, afin de n'aggraver ou de ne créer aucune inégalité. Malheureusement, les récents appels à la grève, provenant pour beaucoup des collèges, et les nombreux témoignages d'enseignants désemparés traduisent bien un ratage de plus dans votre méthode. Le monde éducatif déplore des directives inadaptées, et surtout un total manque de temps pour les mettre en oeuvre. Les chefs d'établissements comme les collectivités n'ont eu parfois que vingt-quatre heures avant la rentrée des vacances de la Toussaint pour se conformer aux nouveaux protocoles sanitaires. Les mesures de distanciation ou le suivi des règles d'hygiène sont difficiles, voire impossibles à appliquer. La présence en alternance des élèves, évoquée pour le lycée, n'est pas envisagée au collège, où pourtant le brassage des élèves est tout aussi important, et les enfants tout aussi contagieux. Le risque de devoir fermer des classes et de devoir renvoyer les élèves chez eux est réel., ce sont eux, et particulièrement les plus défavorisés, qui pâtissent de vos décisions. Dans les quartiers et les zones rurales qui n'offrent pas d'activités périscolaires ou qui manquent de moyens numériques, cela ne fera que creuser les inégalités. À l'impossible nul n'est tenu, monsieur le ministre. Pour assurer cette continuité pédagogique, le recrutement de personnels supplémentaires et de remplacement apparaît comme une évidence, afin de restaurer la confiance entre votre gouvernement et la communauté éducative, et d'éviter ainsi à celle-ci l'épuisement que connaissent actuellement nos équipes soignantes. Pourtant, vous ne l'avez pas envisagé, contrairement à ce qu'ont décidé les collectivités locales, qui une fois de plus sont le dernier rempart face aux défaillances de l'État. aux défaillances de l'État. Monsieur le ministre, faudra-t-il une troisième vague pour que ce Gouvernement mette enfin en oeuvre la concertation que la communauté éducative et les élus attendent ?

moins d'élèves. Oui, nous engageons des moyens supplémentaires, cela se voit aussi dans le budget pour l'année prochaine. Puisque vous avez soutenu d'autres gouvernements dans le passé, je vous rappelle un chiffre : 6 milliards d'euros d'augmentation budgétaire pour l'éducation sous ce quinquennat, contre 2 milliards d'euros sous le quinquennat précédent. Faites la comparaison

question s'adresse à M. le Premier ministre. La laïcité à la française, à laquelle nous sommes tous attachés, a deux versants. Pour le premier, la religion n'a pas à s'immiscer dans les affaires de l'État, conformément à la séparation du spirituel et du temporel ; la loi de 1905 est la loi de séparation des Églises et de l'État. L'autre versant de la laïcité est l'obligation faite à l'État de respecter toutes les croyances et de ne pas intervenir dans les convictions de chacun l'État doit assurer la liberté de culte, qui a rang, dans notre pays, de liberté fondamentale. Votre décision de limiter ce qui est essentiel à la fréquentation des grandes surfaces a restreint cette liberté fondamentale le Conseil d'État, au travers d'une jurisprudence constante, qui s'attache à examiner la proportionnalité de la mesure, a confirmé votre décision ; voilà qui est surprenant En quoi est-il plus dangereux de prendre les transports en commun que de se rendre dans un lieu de culte, où les règles de distanciation sociale peuvent être parfaitement respectées ? Monsieur le Premier ministre, vous avez choisi la technique pour oublier la peur, quitte à priver les croyants de l'indispensable recueillement qu'imposent les traumatismes de la pandémie. Faire autrement n'est qu'une question de volonté, et je sais que vous pouvez le faire. Le Conseil d'État vous a demandé de préciser les conditions dans lesquelles les fidèles ont la possibilité de se rendre individuellement dans un lieu de culte. Peuvent-ils s'y rendre lorsque celui-ci est distant de plus d'un kilomètre ? vous a également enjoint de réexaminer votre décision à la mi-novembre- nous y sommes -en lien avec les représentants des cultes. Expliquez-vous sur les mesures de concertation et d'assouplissement que vous comptez prendre

difficile et éprouvante pour l'ensemble du pays, et qui conduit nécessairement les croyants à vouloir se retrouver, à vouloir se recueillir, à vouloir prier peut-être plus encore. Comment ne pas avoir une pensée pour nos compatriotes catholiques, après l'attentat de Nice ? La situation sanitaire nous a conduits à prendre une décision difficile, celle du confinement, pour limiter les risques de contamination, avec une fermeture des établissements recevant du public, pour des raisons sanitaires, pour protéger tous les Français. Pour autant, parce que nous sommes attachés au respect des libertés, notamment au respect de la liberté de culte, nous avons décidé de maintenir les lieux de culte ouverts

au premier confinement, afin que chacun puisse vivre dignement son deuil. Cette situation reste imparfaite, nous le savons. Le Conseil d'État l'a confirmé. Nous savons que les restrictions sont dures, et croyez bien que notre souhait est qu'elles puissent être levées dès que possible. C'est la raison pour laquelle je peux vous annoncer qu'une réunion se tiendra au ministère de l'intérieur, dès le début de la semaine prochaine, probablement dès lundi prochain, en présence des représentants

dès maintenant, car, dès que cela sera possible, nous avons le souhait de pouvoir permettre aux croyants de rejoindre ces lieux de culte. Nous sommes extrêmement mobilisés, et nous allons construire ces solutions avec les représentants des cultes. Dois-je vous rappeler que sous prétexte d'irrégularités constatées par vidéo sur le respect des consignes sanitaires dans deux diocèses, à savoir Bayonne et la Martinique, le Conseil d'État englobe dans sa décision tous les autres lieux de culte ? Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de cluster déclaré en ces lieux. lieux. Aucun ! Nos concitoyens ont perdu la confiance. C'est dommage, c'est triste ! Ce n'est pas à l'honneur de la République ! Alors ne leur imposez pas de perdre leur espérance !

et Républicain. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Monsieur le ministre, vous disiez la semaine dernière vouloir que la France tienne sa place dans la médiation du conflit en Artsakh. La France et l'Union européenne sont hors-jeu. L'accord signé lundi sous l'égide de la Russie montre notre incapacité à compter. La communauté internationale, en ne s'opposant pas à cette irruption de la force militaire dans un conflit séculaire, renonce dans le mais aussi dans tout le Proche-Orient, à la possibilité d'une gestion diplomatique des conflits et à la protection des droits humains, laissant ainsi les mains libres aux ambitions de M. Erdogan. Ce conflit, dit a trouvé une issue par la force, la violence et la haine. Cette évolution en plein coeur du sud du Caucase est une catastrophe. Plusieurs milliers de jeunes appelés ont trouvé la mort. Jusqu'à 90 000 personnes pourraient être contraintes à l'exode. M. Poutine a déclaré que les termes de l'accord permettent aux personnes déplacées de retourner au Haut-Karabakh, alors que le président Aliev s'est félicité d'avoir « chassé les Arméniens de nos terres comme des chiens ». Dans ces conditions, comment les populations déplacées peuvent-elles y retourner ? Dans le groupe de Minsk, quelle est la place exacte de la France ? Allons-nous continuer à nous cacher derrière notre coprésidence ? Aurions-nous totalement perdu la mémoire et sacrifié nos valeurs de démocratie et de liberté ? Qu'est-ce que votre gouvernement compte faire pour protéger les populations et garantir la stabilité de cette région ? Avons-nous les moyens d'établir la réalité des accusations sur l'usage par l'Azerbaïdjan de bombes à fragmentation et au phosphore ? allez-vous proposer des sanctions face à ces crimes de guerre ?

Il importe qu'il soit respecté. Cette guerre a été meurtrière ; cette guerre a été d'une très grande brutalité ; elle a été dramatique. Les combats ont maintenant cessé, il faut que le cessez-le-feu soit respecté totalement, par toutes les parties. Doivent maintenant s'ouvrir les discussions, sur la base du cessez-le-feu, pour en définir les différents paramètres, pour faire en sorte qu'un vrai règlement du conflit dans le Haut-Karabakh puisse avoir lieu, sur le long terme.

Cette initiative reçoit l'appui des autorités arméniennes. D'ici là, il faut s'assurer non seulement que le cessez-le-feu soit totalement respecté, mais aussi que les combattants étrangers

que l'énorme effort humanitaire que la France veut déployer à l'égard des Arméniens se mette en oeuvre. Les opérations ont déjà commencé ; d'autres initiatives seront prises, vous le constaterez dans l'après-midi, à la suite d'une rencontre au plus haut niveau entre les autorités de l'État français, les ONG et la communauté arménienne

et moyennes entreprises. Monsieur le ministre, l'impact économique et social de la fermeture des établissements qui reçoivent du public et l'interdiction d'organiser tout rassemblement ou événement placent le secteur de l'événementiel dans une situation dramatique. Il s'agit pourtant d'une filière qui est essentielle pour l'attractivité de notre pays, pour l'attractivité des territoires et pour notre secteur touristique. En France, chaque année, sont organisés 1 200 foires et salons, 2 800 congrès et 380 000 événements d'entreprises et d'institutions. Plus de 77 millions de participants sont ainsi accueillis chaque année, dont 10 % de participants d'origine étrangère. Au coeur de la crise se trouvent notamment les traiteurs, organisateurs de réception, qui travaillent avec une clientèle tant de professionnels que de particuliers. Depuis le printemps, plus de 17 000 entreprises sont ainsi à l'arrêt, inquiètes pour leur avenir économique, y compris les entreprises phares du secteur. Je voudrais aussi terminer cette intervention en évoquant le sort des extras, les 70 000 intermittents de la restauration, monsieur le ministre ! Les entrepreneurs de foire, de salons, de congrès,

Par ailleurs, vous nous parlez des traiteurs. J'ai personnellement reçu à sept reprises les représentants des traiteurs, les Traiteurs de France, les Traiteurs de Paris, pour examiner une situation qui est- vous avez raison -très difficile

essentielle pour notre pays, parce que ce sont eux qui nous permettent d'organiser les meilleurs événements.

Le confinement a donc eu pour eux un effet négatif. Nous constatons aussi que les élèves du cycle 2 ont été plus fragilisés que ceux de sixième. Plus âgés, ces derniers sont probablement plus autonomes vis-à-vis des outils de l'école à distance, et moins touchés par une absence de présence à l'école et de contact avec leurs professeurs. Enfin, si le dédoublement des classes de CP et CE1 avait eu un effet positif, la crise l'a clairement annulé. Cela confirme le rôle essentiel du temps personnalisé passé par l'enseignant aux côtés de chaque élève. Les déterminants liés à un environnement socio-économique défavorable sont bien compensés par l'école de la République, encore faut-il qu'elle soit physiquement présente. D'où l'importance du rôle des enseignants et de l'école comme structure sociale et éducative pour effacer les différences. Monsieur le ministre, dès lors, plusieurs questions se posent. Bon nombre d'élèves ont été déscolarisés ou sous-scolarisés pendant et après le confinement. Ont-ils bien tous été identifiés ? Quels moyens avez-vous mis en place pour remédier individuellement à ces effets négatifs ?

Enfin, cette cohorte d'élèves a vécu une expérience inédite aux nombreuses conséquences, sur le plan des acquis et sur le plan psychologique. Va-t-elle faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation spécifiques renforcés dans le temps, tant au niveau pédagogique que par la médecine scolaire ? Je vous remercie.

en souligner l'importance devant l'ensemble des sénateurs et sénatrices. Il s'agit de la situation de l'école primaire, alors même que nous vivons cette crise sanitaire. Dans un contexte mondial, où on ne dira jamais assez qu'une

Monsieur le président, ma question s'adresse à M. le Premier ministre et porte sur la gestion du covid-19. Monsieur le Premier ministre, vous êtes encore appelé, ce soir, à annoncer des mesures qui portent atteinte, d'une manière inédite en temps de paix, à nos libertés fondamentales. Si, dans son principe, le Parlement a parfaitement admis, quoi que vous en disiez, la nécessité d'une action rapide en la matière, une difficulté majeure se pose quant à la proportionnalité et à la justification des mesures ainsi adoptées. En effet, vous disposez de nombreuses informations

fleurs ou des jouets, les salons de coiffure et tant d'autres sont quinze fois moins dangereux que d'autres catégories de commerce, ce qui tend à prouver une certaine forme d'inutilité de vos choix hétéroclites pris dans l'urgence, sous la pression d'un virus qui mène la danse.

le contrôle du Parlement, Assemblée nationale comme Sénat, a été constant depuis le début de cette crise à travers l'ensemble des outils dont les

en application de cet état d'urgence. Ensuite, sur la question de la concertation et de la coopération avec les

à quel point une telle décision peut altérer la continuité d'activité de ce site. Le Gouvernement est parfaitement conscient de la nécessité d'agir pour assurer cette continuité, mais, vous le savez, le recrutement et la formation de nouveaux agents peuvent prendre entre six mois et un an. Or nous n'avons pas le temps d'attendre. C'est la raison pour laquelle, afin de pallier toute difficulté, l'établissement

tant la situation est tendue dans nos hôpitaux. La deuxième vague est là. Nos personnels soignants sont sur le front. Nos concitoyens font preuve de civisme et respectent très majoritairement les mesures visant à limiter la propagation du coronavirus. Cependant, nous vous entendons très peu sur la prise en compte des conséquences humaines de ces périodes de confinement. Une bonne santé mentale permet aux personnes de mieux surmonter les tensions normales de la vie, mais en cette période de crise sanitaire, nous sommes confrontés à une situation anormale. Contraindre toute une population à limiter pendant plusieurs semaines tous ses contacts pas de les interdire, a inévitablement un impact néfaste sur la santé mentale de tous. Les Français ont subi un premier confinement qui a laissé des traces stress, ennui, frustration, perte inédite de liberté, isolement, peur de tomber malade, baisse de l'activité physique ont déjà laissé des séquelles qui risquent encore de s'aggraver. Avez-vous répertorié précisément ces troubles ? Pouvez-vous porter à notre connaissance une analyse précise de l'état mental de la population ? Beaucoup de Français vous reprochent de ne pas bien gérer l'après-confinement. Les annonces, souvent contradictoires, ont elles aussi suscité de l'angoisse et un manque de confiance chez nos concitoyens. Gouverner, c'est prévoir. Et pour prévoir, il faut connaître exactement l'évolution de l'épidémie, certes, mais aussi les impacts psychiques sur la population. Monsieur le ministre, le premier confinement était une expérience. Il a eu lieu il y a plus de cinq mois.

Une autre enquête récente de Santé publique France révèle, chez nos concitoyens, une augmentation de plus de cinq points des troubles dépressifs en octobre par rapport au mois précédent, avec une persistance des troubles du sommeil.

Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Compte tenu de la situation très inquiétante dans laquelle se trouvent aujourd'hui nos hôpitaux, j'ai approuvé la décision prise par le Gouvernement de procéder à un nouveau confinement, malgré les conséquences pour nos entreprises.

le pire serait que le futur déconfinement, que nous attendons tous, connaisse les mêmes errements que le premier- je pense notamment à l'absence d'obligation de porter un masque que rien ne pouvait justifier. Nos entreprises, nos commerçants devront une nouvelle fois improviser et découvrir le dispositif au dernier moment, dans la confusion et l'urgence, sans avoir le temps de s'y préparer. Nous avons besoin d'une stratégie de déconfinement précise et connue de tous à l'avance, d'un protocole clair avec des interlocuteurs Le protocole d'ouverture d'un salon de coiffure ou d'un restaurant ne peut pas être pensé comme celui d'une librairie ou d'une salle de sport. Monsieur le Premier ministre, ce que nous voulons- c'est le restaurateur qui vous parle -, c'est travailler ! Nous sommes en train de perdre notre patrimoine, notre retraite. Nous ne voulons pas être sous perfusion, même si nous avons bien sûr besoin des aides de l'État ; nous voulons surtout travailler et faire travailler nos collaborateurs dans le respect des règles sanitaires et de la santé de chacun. Donnez-nous des perspectives ! Une concertation entre les préfets, les maires, les forces vives du territoire et les soignants doit permettre, dès à présent, d'ajuster localement les protocoles. Il faut un déconfinement sur mesure. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous en mesure de nous apporter des assurances en termes de calendrier pour anticiper ces protocoles localisés et d'engagement de l'État sur une communication claire et accessible en direction des acteurs concernés ? La

comme à nous, doit être de tout mettre en oeuvre pour que notre système sanitaire tienne bon. C'est ce à quoi nous nous employons depuis le début de cette crise et c'est tout le sens des mesures que nous prenons : augmentation progressive des capacités en réanimation, formation

Le suivi épidémiologique et sanitaire est un élément essentiel pour analyser l'évolution des contaminations. Il faut conclure ! Ce suivi se poursuit sur tout le territoire grâce à l'action de milliers d'hommes et de femmes que je salue ici et je vous garantis, monsieur le sénateur, que ce soir nous serons en mesure de dresser les perspectives, en fonction de la situation sanitaire

J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sien de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein

L'article 14 a pour objet de permettre aux particuliers réalisant des activités économiques sur les plateformes numériques de bénéficier d'un dispositif social ultra-simplifié : cotiser en s'inscrivant sur un service en ligne unique, sans aucune formalité, dès lors que l'activité produit des recettes annuelles inférieures à 1 500 euros.

Ces activités présentent potentiellement un risque important d'accidentologie, qui nécessite un exercice professionnel et une prévention des risques professionnels adaptés. Nous proposons donc

partie. Il s'agit de permettre à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de prendre des mesures conservatoires, évidemment préventives,

redressement-recouvrement, qui est identique en matière de fraude fiscale, est totalement dépassé lorsque les sociétés contrôlées organisent leur insolvabilité soit sur une liquidation soit en cas d'engagement de contrôle. C'est aussi le cas des entreprises éphémères.

du Gouvernement ?

Cet amendement, à la différence du précédent, avait été adopté l'année dernière, mais sa durée de vie avait été un peu identique

2020. Il s'agit de clarifier la caractérisation comme outil professionnel de la carte accordée par nécessité de service aux 55 000 salariés relevant de la convention collective nationale du transport urbain. Cela concerne tous les opérateurs de transports publics. Pendant près de dix ans, et jusqu'à récemment, toutes les caisses d'Urssaf ont systématiquement assimilé la carte de service à un outil de travail en suivant une doctrine basée sur le droit social et la réalité d'usage de celle-ci. Or certains contrôles se sont récemment

été débattu l'an dernier. M. Dussopt nous avait indiqué que l'évaluation de ce qui relevait d'un avantage devant être assujetti à cotisation était complexe. On n'en doute pas

cependant que cet amendement avait été voté à l'unanimité l'année dernière. Il a été redéposé, parce que la négociation avec l'Acoss, qui aurait pu être une solution,

Monsieur le rapporteur

Cet amendement vise à mettre fin à la distorsion de concurrence entre les professionnels de la location de biens meublés selon qu'ils passent par des plateformes numériques d'échange de biens ou non. ou non. Nous proposons de clarifier le cadre social applicable aux loueurs professionnels louant des biens meublés sur ces plateformes en faisant contribuer à la solidarité sociale nationale les professionnels du tourisme qui les utilisent au même titre que les acteurs de l'économie traditionnelle.

En effet, un loueur louant sa résidence principale jusqu'au seuil maximum de 120 jours par an à un prix moyen de 80 euros la nuit peut gagner jusqu'à 9 600 euros par an sans que ces revenus soient soumis au moindre euro de cotisation sociale. En revanche, les loueurs de biens dits meubles, comme des voitures ou des tondeuses, sont assujettis aux cotisations sociales dès le dépassement du seuil de 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 8 104,80 euros en 2019.

Il s'agit ainsi de faciliter le contrôle de l'activité de location de locaux d'habitation meublés à titre lucratif. Dans son principe, une telle mesure est similaire à l'obligation de déclaration auprès du fisc qui figure dans la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Nous souhaitons faire en sorte que ces plateformes transmettent systématiquement aux Urssaf les informations collectées sur les revenus issus des locations de biens meublés. Les plateformes de mise en relation deviendraient ainsi des tiers déclarants, comme peuvent déjà l'être aujourd'hui les associations et centres de gestion ou les cabinets d'expertise comptable, la déclaration sociale nominative. Elles seraient également chargées du versement des cotisations et des contributions sociales. En règle générale, nous sommes particulièrement vigilants à l'égard des disparités de traitement entre les plateformes et les acteurs du commerce plus traditionnel, qui subissent encore aujourd'hui le manque d'adaptation de la loi à ces nouvelles formes de concurrence. Il s'agit d'un amendement de bon sens, qui permet de clarifier la transmission des informations et de limiter la fraude, combat cher à notre Haute Assemblée. Très

tout sens et aboutit à ce que les plateformes réalisent elles-mêmes la déclaration et le paiement des cotisations. Le II vise à prévoir la transmission par les plateformes des données concernant, notamment, l'utilisateur et les transactions réalisées,

Monsieur le ministre, fiscales et douanières, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, de collecter et d'exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateformes pour faciliter la recherche des infractions graves à la réglementation fiscale et douanière. Un rapport

sont insupportables pour le plus grand nombre de nos concitoyens. Ils voient bien que de grandes entreprises touchent des aides publiques et licencient, qu'elles continuent de bénéficier des plans d'aide, comme Amazon,

de la fraude sociale provient des mauvaises déclarations, intentionnelles ou non- quand il s'agit de fraude, c'est intentionnel -des entreprises qui sous-estiment leurs versements de cotisations.

cet article rétablit l'attribution au contentieux général de la sécurité sociale des litiges susceptibles de naître lors du recouvrement de la contribution liée à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, qui finance

le prétexte suivant : « L'utilisation de procédures dématérialisées n'est jamais une obligation ; il existe toujours des moyens matériels d'accéder aux services publics. » L'article 15, dans sa formulation actuelle, vient contredire ce principe, mais aussi les préconisations exprimées par le Défenseur des droits dans son rapport de 2019

En application de l'article 1649 B du code général des impôts, les professionnels non salariés, comme les exploitants agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles, sont d'ores et déjà soumis à une obligation de dématérialisation pour la déclaration de leurs revenus fiscaux professionnels,

À ce jour, seule la déclaration fiscale personnelle de revenus ne fait pas encore l'objet d'une obligation généralisée de dématérialisation, compte tenu des difficultés rencontrées par certains déclarants. Toutefois, il est important de rappeler que la possibilité d'effectuer cette déclaration sur papier prendra fin pour

Monsieur le ministre,

rapporteur général. Cet amendement vise à limiter la possibilité laissée aux organismes de sécurité sociale de moduler les annulations de réductions de cotisations lorsque le travail dissimulé reste très réduit. d'interdire toute possibilité de moduler la sanction lorsque l'infraction est commise en bande organisée et de préciser que le plafond de l'activité dissimulée permettant la modulation est le même quel que soit le nombre de salariés concernés.

de cotisations vieillesse concerne seulement les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité (Sicae), et non l'ensemble des salariés des industries électriques et gazières

correspondant au versement des salaires. En cas de fraude, les entreprises doivent immédiatement remplir ou corriger toutes les déclarations manquantes. L'amendement est donc sans effet sur ce point. De manière générale, nous n'avons pas intérêt à empêcher les entreprises à risque de fraude de réaliser des déclarations selon les modalités habituelles. L'objectif est plutôt qu'elles les remplissent, pas que chaque organisme reçoive des informations séparées

pour les sphères fiscales et sociales. La règle la plus favorable aux redevables est toujours d'imputer d'abord les versements sur les dettes dues à titre principal pouvant faire courir des intérêts et des pénalités de retard.

présenté par M. Jomier,

contre le non-recours aux prestations sociales, déjà en temps normal et plus encore en cette période de crise, dont vous avez rappelé qu'elle affectait au premier chef les plus modestes de nos concitoyens.

CAF à travers les rendez-vous des droits, qui sont proposés aux allocataires et qui permettent d'étudier leur éligibilité aux différentes prestations sociales. Par ailleurs, le portail numérique, à défaut de résoudre de résoudre toutes les situations, contribue aussi à informer les allocataires et à leur permettre de simuler leurs droits à de nombreuses prestations. Ces rendez-vous des droits se multiplient dans les territoires au sein des différentes CAF.

Les échanges d'informations entre les organismes seront ainsi autorisés pour détecter, par des techniques dites de, les personnes éligibles aux différentes prestations et les informer de leurs droits, afin qu'elles puissent en faire la demande.

à mettre en place un tel dispositif pouvant créer des effets de bord contreproductifs, et vous allez être amenés à améliorer les dispositifs existants, notamment en permettant aux organismes de sécurité sociale de s'attaquer au problème

Si l'État ne s'impose rien à lui-même en matière de droits devant être garantis aux plus fragiles, il n'est pas à la hauteur de l'espérance républicaine

qui leur sont nécessaires pour apprécier si un allocataire a droit à une prestation et pour la lui proposer.

et affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale français, ayant souvent accompli une partie de leur carrière en France. Contrairement aux retraités résidant en France, ils ne sont pas assujettis

en contrepartie de laquelle leur est garanti l'accès aux services de la sécurité sociale en cas de séjour ou de retour en France. Les pensions de base sont actuellement

Vous souhaitez appliquer cette progressivité en fonction du revenu fiscal de référence des personnes concernées, comme cela est le cas pour la CSG acquittée par les résidents. Toutefois, par définition, ces personnes ne disposent pas d'un revenu fiscal de dans la mesure où elles n'ont pas leur résidence fiscale en France. Il serait donc impossible d'appliquer un tel barème. En effet, même si certaines d'entre elles déclarent une partie de leurs revenus en France, cela ne permet pas d'apprécier l'ensemble de la capacité contributive des titulaires des revenus de remplacement. Dès lors, le montant total de leurs revenus est inconnu. Par ailleurs, il ne paraît pas non plus possible d'introduire une forme de progressivité sur leur pension de source française, car, même si ses revenus sont connus, ils ne constituent là encore qu'une partie de leurs ressources. Il n'est pas certain

Par conséquent, même si cette cotisation n'est pas progressive, elle ne peut pas être comparée avec la CSG, et elle reste dans la quasi-totalité des cas beaucoup plus faible que la CSG prélevée sur les résidents.

Dans son rapport sur la mobilité internationale des Français, la députée de la onzi circonscription des Français établis hors de France, Anne Genetet, propose de modifier le code de la sécurité sociale en vue de permettre la prise en charge des conjoints dont les frais de santé ne sont pas couverts par le droit européen ou international. Dans la mesure où, au regard de l'article 40 de la Constitution, le Parlement n'a pas la possibilité d'élargir le champ d'application du code de la sécurité sociale, en sorte que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant la possibilité de concrétiser la proposition formulée par Mme Genetet. Quel est l'avis de la commission ?

l'avis du Gouvernement ?

pour des soins en France. Le sujet a fait l'objet d'une instruction ministérielle au mois de juillet 2019 visant à faciliter la transition pour les personnes concernées. L'équilibre trouvé à l'époque nous semble le bon. Nous ne souhaitons pas revenir dessus. Le Gouvernement émet

une meilleure équité territoriale dans l'offre d'accompagnement. En effet, certains départements ruraux ayant une proportion de personnes âgées dépendantes très importante seront confrontés à des problèmes économiques, notamment avec une augmentation des personnes accédant au RSA, et à de graves soucis financiers pour prendre correctement en charge la dépendance en établissement et à domicile. Cette branche intègre aussi l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Nous sommes donc parfaitement en phase avec les objectifs de la loi.

mais au moins rapidement passer de 0,3 ETP à 0,4 ETP. Le financement de l'économie dans le texte est de 31 milliards d'euros. Il est en fait l'addition du regroupement des financements de 2019 et de l'augmentation des salaires du Ségur de la santé, que je salue.

L'attractivité des métiers d'aides-soignants et d'infirmiers en Ehpad, c'est le salaire, mais aussi un nombre suffisant de personnels pour pouvoir dialoguer un peu avec les résidents et prendre en charge correctement les pensionnaires très dépendants avec un GMP moyen à 750.

Nous allons discuter de la cinquième branche de la sécurité sociale, chargée de l'autonomie, mesure annoncée comme un marqueur de ce PLFSS. Le groupe SER a acté la création de cette branche l'été dernier, est adossée au transfert de la dette covid aux organismes de la sécurité sociale. À l'époque, le rapport confié à M. Laurent Vachey promettait de répondre aux nombreuses questions subsistantes, et ce avant l'automne. Nous y sommes. Si une intention a été clarifiée, les interrogations subsistent. Ce qui est plus clair, c'est que cette branche autonomie doit s'adresser à toutes les personnes en situation de dépendance, quelle que soit l'origine quelle que soit l'origine : vieillissement ou handicap. Cette incertitude levée- et c'est tant mieux -, il faudra remettre plusieurs fois l'ouvrage sur le métier pour achever la convergence des politiques de prise en charge de l'âge et du handicap. Nous veillerons à encourager la portée universaliste de la prise en charge au travers d'amendements. Nous le savons, la barrière d'âge à 60 ans crée des inégalités de traitement que plus rien ne justifie. Au-delà du périmètre de la branche, les enjeux résident dans son mode de gestion et son besoin de financement. Outre les transferts de CSG, fiscalité proportionnelle, aucune ressource n'est mobilisée pour assurer l'équilibre de cette branche et répondre aux besoins à venir. Nous proposerons donc de faire contribuer les revenus du capital et les successions, tout comme nous veillerons aussi à diminuer le reste à charge des assurés.

consacrés à l'autonomie au sein de la sécurité sociale ; la gestion en sera confiée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. Le rapport Vachey formulait des propositions de financement de la branche perte d'autonomie, dont certaines étaient très dangereuses,

Nous regrettons que le PLFSS entérine la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale financée uniquement par l'impôt. Cette cinquième branche est une nouvelle étape vers une étatisation de la sécurité sociale- c'est d'ailleurs le cas dans les pays anglo-saxons -, qui n'assure qu'un minimum pour les plus précaires et ouvre la porte aux assurances privées. Le financement par une ponction de la contribution sociale généralisée va renforcer la confusion des comptes de la sécurité sociale et de l'État. Même si la prise en charge actuelle de la perte d'autonomie n'est pas acceptable, la réforme proposée va aggraver les injustices. Pour nous, la perte d'autonomie en soi n'est en rien un risque ; c'est un aléa de la vie qui justifie une prise en charge par le régime général de l'assurance maladie, et non par une branche spécifique, comme le propose le Gouvernement.

notamment pour les assurances privées. Nous proposons donc à l'inverse de mettre à contribution les revenus financiers, les dividendes, pour financer une prise en charge de l'autonomie assurée à 100 % par l'assurance maladie.

La manière de délivrer des prestations nouvelles n'est pas encore définie. C'est la raison pour laquelle nous sommes tout à fait favorables à l'avancement du dispositif,

à l'augmentation des traitements du personnel dans les Ehpad. C'est bien- c'était nécessaire -, mais cela ne résout pas le problème du manque évident de personnel dans ces établissements. J'étais tout à l'heure avec un collectif de médecins du CHU de Saint-Étienne.

en plus de pratiquer des tarifs prohibitifs, accueillent les personnes âgées dans des conditions dignes, ce qui n'a pas été le cas, on l'a vu, l'été dernier ? Ce sont des questions étendues sur lesquelles nous attendons des réponses. Nous souhaitons participer au débat.

Donc, on ne fait pas ce qu'on pourrait et devrait faire, et on crée une illusoire cinquième branche qui sert en quelque sorte de paravent à une forme d'impuissance collective.

Cet article ne prend pas du tout en compte la globalité du problème et surtout l'embauche des personnels, leur salaire, la reconnaissance de leur formation et leur accompagnement.

car vous estimez que le risque lié à la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap doit être couvert par l'assurance maladie. Comme l'a rappelé le rapporteur, la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie a affirmé

L'ambition de cette cinquième branche est d'assurer une meilleure équité territoriale dans l'accès aux droits des personnes âgées et des personnes handicapées, d'améliorer l'offre d'accompagnement à destination de ces publics et de renforcer les politiques transversales du handicap et du grand âge. C'est une nécessité. Elle porte également en elle une promesse de démocratie, démocratie, puisqu'à compter de cette année, un examen annuel de la politique de l'autonomie et de son financement à long terme sera opéré dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. Je pense que, là aussi, les parlementaires que vous êtes ne peuvent que s'en réjouir. L'article 16 du PLFSS 2021 tire donc les conséquences de ces évolutions nécessaires. Il vise à organiser le fonctionnement de cette nouvelle branche et à en garantir un financement autonome équilibré. C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à sa suppression.

En l'occurrence, nous considérons que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie doit avoir pour vocation de garantir l'égalité des droits, et non pas simplement un juste traitement.

qui ne correspond ni à notre histoire, encore moins à celle de la création de la sécurité sociale par le Conseil national de la Résistance, ni même à l'affirmation de la promesse républicaine, dont chacun est conscient aujourd'hui qu'il faut lui redonner toute sa force.

Monsieur le ministre, de préciser l'importance, je pense que nous sommes d'accord sur l'objectif. Nous souhaitons, comme vous, que les personnes en perte d'autonomie bénéficient du même niveau de prestations lorsqu'elles se trouvent dans des situations

-visant à renforcer le rôle de la CNSA en matière d'équité territoriale. Nous avons également déposé un amendement tendant à préciser la mission de la CNSA en matière de soutien aux

pour l'autonomie, la CNSA, ont été clarifiées, afin de réaffirmer son rôle, notamment en termes de gestion et de financement du risque, de pilotage, d'animation et d'appui aux différents acteurs des politiques de soutien à l'autonomie. Dans ce cadre, le rôle d'appui et d'accompagnement de la CNSA auprès des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l'autonomie, chargées de l'évaluation et de l'ouverture des droits aux prestations, doit être réaffirmé, en particulier s'agissant de la qualité de service et de l'équité de traitement. Les

de renforcer le rôle des universités dans la formation des professionnels de l'autonomie. L'implication de l'université, garante de la formation tant initiale que continue, semble essentielle dans le rôle de la formation des professionnels de l'autonomie. De plus, les besoins de formation de ces professionnels sont particulièrement centrés sur la coordination entre professionnels, afin de permettre une véritable prise en charge interprofessionnelle autour du patient. Les différentes évolutions récentes des structures de coordination ont complexifié la lecture du maillage territorial pour les professionnels de terrain. Ce n'est notamment que par une formation adaptée que ceux-ci pourront s'emparer de tels outils. La parole est à Mme

Contrairement à ce qui est indiqué dans leur objet, ils ne renforcent pas le rôle de l'université dans la formation des professionnels de l'autonomie. Ils tendent simplement à indiquer que la CNSA exerce sa mission en lien avec les universités. Il ne semble pas utile de lister toutes les entités avec lesquelles la CNSA doit juger bon d'exercer sa mission. L'avis est donc défavorable. L'amendement n° 1012 vise à préciser que la CNSA joue un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie et évalue leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. La CNSA, pour l'heure, finance les MDPH et labellise leur transformation en MDA. L'article 16 ne reprend explicitement que les dispositions relatives au financement des MDPH. Son rôle à leur égard pourrait donc être précisé et, éventuellement, complété. Cet amendement constitue un premier pas. Nous y sommes donc favorables.

universités. La CNSA est d'ores et déjà chargée de contribuer à l'attractivité des métiers, en particulier par ses actions en faveur de la formation et de la professionnalisation. Un amendement a été adopté à cet effet en première lecture à l'Assemblée nationale.

mais l'inscrire dans la loi sans en tirer de conséquences opérationnelles me semble un peu prématuré. Voyons plutôt cela à l'occasion des débats de fond qui se tiendront plus opportunément lors de l'examen de la loi sur le grand âge, et demandons un calendrier

Cet amendement vise à confier à la CNSA la mission d'assurer le libre accès aux prestations d'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il tend également à demander à la CNSA de rechercher des solutions innovantes pour réduire le reste à charge des assurés en matière de dépendance et de perte d'autonomie. Les rapports Libault et El Khomri font état d'un besoin de financement important pour l'autonomie, s'élevant à 6 milliards d'euros par an à partir de 2024, et évoquent des restes à charge substantiels. Aussi, il apparaît nécessaire de donner mission à la CNSA de rechercher des solutions, afin d'améliorer l'accès aux prestations d'autonomie pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

La mission de veiller à garantir l'accès aux prestations n'est pas très précise ; elle et sans doute incluse dans la mission d'information prévue à l'alinéa 7. La mission de contribuer à la recherche d'innovations est déjà prévue à l'alinéa 8. En conséquence, la commission sollicite le retrait l'avis du Gouvernement ?

Ce nouveau service public est particulièrement attendu par les bénéficiaires potentiels, qui auront sans nul doute besoin d'un accompagnement personnalisé pour accomplir leurs démarches. N'oublions pas que la CNSA s'adresse en particulier à des personnes fragilisées, peu mobiles pour certaines du fait de leur handicap et pas très au fait des procédures dématérialisées pour d'autres. Aussi, cet amendement, déposé par mon collègue Jean-Yves Roux, vise à préciser à l'alinéa 7 que des permanences physiques pourront être prévues de droit dans les maisons France Services, en complément des procédures numériques et d'un guichet départemental. Les auteurs de l'amendement insistent par ailleurs sur le fait que ces permanences peuvent aussi donner lieu à des formations aux procédures dématérialisées. Ils mettent en avant la nécessité de prévoir un accès renforcé pour les différentes situations de handicap, que ce soit des déficits visuels et auditifs ou des difficultés de mobilité.

Il est un peu prématuré, et sans doute pas de niveau législatif, de prévoir avec ce niveau de détails la mise en oeuvre de la mission d'information de la CNSA, en anticipant sur les débats qu'ouvrira la loi relative au grand âge et à l'autonomie.

relève des conseils départementaux, les MDPH. La CNSA contractualise avec les conseils départementaux. La feuille de route MDPH 2022 témoigne de sa volonté d'investir massivement dans l'information des bénéficiaires et des familles, mais la CNSA ne peut pas se substituer aux départements pour assurer directement cette information. C'est pourquoi l'avis

bien entendu favorables au principe du guichet unique pour faciliter les démarches des usagers et simplifier le rapport à l'administration. Mais l'insertion

qui sont déjà des structures d'accueil, d'information, de conseil, d'orientation et, le cas échéant, d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; la notion d'autonomie fera

? Cet amendement vise à supprimer la précision ajoutée à l'Assemblée nationale par laquelle la CNSA favorise la création du guichet unique au niveau départemental. Les auteurs de l'amendement craignent que de tels guichets ne concurrencent les structures existantes.

pose les premiers jalons d'un service commun d'instruction des aides aux personnes handicapées ou âgées. Les maisons de l'autonomie, qui n'existent pour l'instant que dans vingt-cinq départements, n'ont pas encore toutes les outils souhaitables, notamment en termes de personnalité juridique, pour devenir le guichet unique de l'accès aux droits et prestations qui seront regroupés dans la cinquième branche. la disposition que vous souhaitez supprimer est au contraire de rendre possible, après une démarche de réflexion et de concertation, une généralisation progressive et un renforcement de ces guichets uniques. C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

actuellement une hausse des demandes de détachement vers la fonction publique hospitalière, mais aussi vers les établissements privés associatifs. Le constat est clair : le statut de fonctionnaire territorial ne semble plus suffisamment attractif et valorisé. Certains agents choisissent même d'abandonner leur statut de fonctionnaire pour aller travailler dans les établissements privés associatifs. Avec le maintien du concours de la fonction publique territoriale pour les personnels, le risque est grand de voir

Dans les Ehpad territoriaux, les agents sont obligés de passer un concours pour pouvoir être titularisés, alors qu'au sein de la fonction publique hospitalière, le personnel est titularisé ou peut bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Plus généralement, nous notons à l'heure actuelle que les instituts de formation des aides-soignants ne séduisent plus. Après le concours d'entrée, les promotions sont incomplètes et beaucoup d'apprenants abandonnent dès les premiers mois d'enseignement. Nous proposons donc d'inscrire dans la loi le principe d'une évolution prochaine des modalités de recrutement au sein de la fonction publique territoriale, en vue d'obtenir à terme une meilleure reconnaissance et valorisation des métiers.

L'idée est intéressante, mais une telle précision n'est sans doute pas à sa place dans un alinéa relatif à l'information des personnes en perte d'autonomie

un certain nombre d'amendements visent à diversifier les missions de la CNSA pour renforcer son rôle d'acteur territorial de l'autonomie. C'est une bonne chose, mais la question de l'assouplissement des conditions d'accès

dans une logique de « parcours » qui permet d'éviter les situations de rupture et de réduire les inégalités. Avant la crise sanitaire, la stratégie de prévention de la perte d'autonomie pour vieillir en bonne santé, présentée le 16 janvier 2020, avait retenu la lutte contre l'isolement comme un élément à part entière de la prévention de la perte d'autonomie.

de la CNSA sur deux points : la promotion des métiers participant à l'accompagnement et au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et la prévention et la lutte contre l'isolement de ces personnes. Les trois amendements suivants

les missions de prévention et de lutte contre l'isolement. C'est aussi l'objet d'un travail que nous sommes en train de réaliser avec mon collègue Bernard Bonne et que nous remettrons prochainement à Mme la ministre Brigitte Les éléments ont été donnés. En regardant de près, j'ai l'impression qu'ils sont presque satisfaits : nous avons voté l'amendement n° 401 rectifié, qui portait aussi sur ces thématiques de lutte contre l'isolement et de prévention de la perte d'autonomie.

de l'autonomie. Il vise à réaffirmer l'importance de la prévention, partie intégrante d'un accompagnement global dans une logique dite de parcours, pour éviter les situations de rupture et réduire les inégalités. Dans le champ des personnes âgées- c'est tout l'intérêt de cette branche autonomie, qui va aligner les personnes âgées dans un même mouvement avec les personnes en situation de handicap -et

La précision trouverait peut-être mieux sa place dans la convention d'objectifs et de gestion que dans la loi. Au regard de l'enjeu, je demande l'avis du Gouvernement. ? Madame la sénatrice, vous demandez que la CNSA introduise dans ses réflexions prospectives sur les politiques de l'autonomie leurs possibles adaptations territoriales. La rédaction proposée des missions de la CNSA prévoit d'ores et déjà qu'elle prend en compte les spécificités de tous les territoires et ne la limite pas dans ses réflexions prospectives. lui permet de proposer, le cas échéant, des adaptations territoriales. La CNSA développe activement des actions d'accompagnement spécifiques aux régions, collectivités ou territoires d'outre-mer, pour répondre déjà leurs besoins. Je partage la nécessité d'apporter une réponse adaptée à chaque situation en tenant compte du contexte spécifique et des besoins d'autonomie de la personne. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait que nous partageons la même ambition, j'émets un avis de sagesse.

le recours à des prestations extérieures est plus rapide. C'est l'inverse lorsque la femme aide son partenaire. La politique de prévention que nous souhaitons confier à la CNSA devrait idéalement s'intéresser aux différences de genre et considérer les inégalités liées au sexe, afin d'élaborer des mesures correctives. Quel est l'avis de la commission commission ? Il s'agit de préciser que la réflexion prospective de la CNSA prend en considération les inégalités liées au sexe afin d'élaborer des mesures correctives. C'est un aspect important,

structures d'accompagnement des personnes âgées dans le champ médico-social ont vu le jour ces dernières années. Celles-ci, tout en permettant d'offrir un meilleur soutien à cette population, ont complexifié la lecture du maillage territorial

regroupant l'ensemble des acteurs, afin de limiter le fonctionnement en silo. Ces structures, nommées maisons des aînés et des aidants, existent déjà sur certains territoires. Cet amendement vise à confier à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie la responsabilité d'en définir le champ et d'accompagner leur développement sur le territoire.

À l'instar des précisions sur le rôle des maisons départementales de l'autonomie, il est sans doute un peu tôt pour préciser dans le budget de la sécurité sociale le maillage territorial fin des guichets d'information en matière d'autonomie, qui fera l'objet de débats lors de l'examen de la loi grand âge.

en assurant l'association des représentants d'usagers dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées à l'échelon local. Il est indispensable que les usagers puissent contribuer aux côtés des professionnels aux travaux liés au soutien à l'autonomie, à l'accompagnement de la dépendance et du handicap. Par ailleurs, pour que la démocratie médico-sociale soit particulièrement vivante, il est nécessaire de favoriser l'essor des réseaux associatifs sur l'ensemble des territoires. Quel

du Gouvernement ? Madame la sénatrice, je soutiens pleinement la démocratie médico-sociale et la représentation des usagers dans les instances nationales ou locales. Cette démocratie existe déjà l'échelon régional, avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, et à l'échelon départemental, avec les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, créés par la loi de 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et dont le premier collège représente des usagers : personnes handicapées, personnes âgées et aidants. La participation des usagers est recherchée dans le champ médico-social. Ainsi la Haute Autorité de santé mène-t-elle une enquête de grande ampleur auprès des usagers du secteur. Cependant, les évolutions à apporter pour favoriser l'essor de la démocratie médico-sociale relèvent du domaine de la loi, et non des orientations données par une caisse de sécurité sociale. C'est pourquoi, tout en partageant votre ambition, j'émets un avis défavorable sur votre amendement.

On est encore dans une série de sigles qui montre bien que l'articulation est difficile dans ce secteur ! Laissons donc faire les territoires. N'en rajoutons pas. Ils s'organiseront par eux-mêmes. Ce sera beaucoup plus efficace. Je mets

pour la cinquième branche autonomie, alors que le présent projet de loi n'est pas à la hauteur des besoins de financement identifiés par le rapport Libault de mars 2019, à savoir 6,5 milliards d'euros en 2024. Alors que l'encours des produits d'assurance vie représentait plus de 1 800 milliards d'euros début 2020, même une faible mobilisation de ces réserves permettrait d'obtenir un rendement intéressant, de l'ordre de 2 milliards d'euros. Le présent amendement vise donc à mettre en place un prélèvement exceptionnel de 0,5 % sur ces encours. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux personnes physiques ayant des encours d'assurance vie supérieurs ou égaux à 100 000 euros. Quel

l'avis du Gouvernement ?

d'euros à l'investissement dans l'immobilier, l'équipement et le numérique en faveur du médico-social. Enfin, un ensemble de mesures en faveur du handicap viennent traduire les engagements de la Conférence nationale du handicap pilotée par Mme la secrétaire d'État. Pour financer une grande partie de ces dispositifs, la CNSA bénéficie désormais, à compter de ce PLFSS, d'un financement autonome grâce à des recettes propres. En tout, ce sont 28 milliards d'euros de CSG qui seront déjà affectés à la branche. Au total, vous le savez, la branche autonomie représente des dépenses à hauteur de 31 milliards d'euros. Bien entendu, tout cela n'épuise pas

Vachey, qui vous a été remis mi-septembre, rapport aussi riche qu'exhaustif. Vous le savez, l'équation est difficile. Entre les transferts, les économies et les nouveaux prélèvements obligatoires, la voie de passage n'est pas simple. Elle l'est peut-être encore moins aujourd'hui, en période de crise.

vous vous y engagez, et j'en suis ravie, car cela fait plus de deux ans que c'est reporté. L'autonomie subit des reports dilatoires ; ce n'est jamais le moment.

vous ne pourrez rien faire pour améliorer l'attractivité des métiers du prendre soin dès l'année prochaine : vous allez donc encore sinistrer davantage le secteur. Autrement, si vous voulez

conscientes que ces annonces ne seraient pas perçues favorablement par l'opinion. Les pouvoirs publics et les organisations professionnelles ont multiplié les appels à la modération. Le gouvernement français a consenti à faire du non-versement des dividendes et de rachat d'actions une condition pour bénéficier d'un prêt garanti de l'État ou d'un report de cotisations, mais pas pour bénéficier du chômage partiel ou de l'appui des banques centrales. Au final, un petit tiers du CAC 40 a annulé ou suspendu le versement des dividendes initialement prévu, essentiellement les grandes banques, qui ont été indirectement obligées de pouvoir avoir accès au refinancement bancaire la Banque centrale européenne, la BCE, ainsi que de grands groupes ayant un urgent besoin d'aides publiques pour survivre à la période. Plusieurs n'ont pas totalement abandonné l'idée de verser un dividende un dividende plus tard dans l'année. Au final, au titre de l'exercice 2019, les actionnaires ont reçu 34 milliards d'euros alors même que la pandémie sévissait, que l'économie était à l'arrêt et que des millions de salariés étaient placés en chômage partiel. Alors que le vieillissement de la société impose de dégager de nouvelles recettes pour la sécurité sociale, nous proposons que la branche « perte d'autonomie » bénéficie d'une contribution des dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 2 %. Cette mesure permettrait

Cela pose-t-il problème ? Pas nécessairement, mais cela interroge surtout au regard des besoins futurs. Nul doute que la sécurité sociale aura du mal à résister aux transferts toujours plus importants de la CSG vers la branche d'autonomie dans les années à venir. Cet amendement vise à prévoir un élément supplémentaire dans le financement de la branche. Ces nouvelles ressources- j'insiste sur ce point -viendront en déduction de la part de CSG transférée à la CNSA. Le Gouvernement et notre rapporteur général devraient y voir un moyen de participer au rétablissement des comptes de la sécurité sociale.

Sur le droit de propriété, la CDC est dépositaire des fonds et doit donc les rendre quand on les lui réclame, comme une banque. Cela n'empêche cependant pas nos banques d'utiliser notre argent pour des opérations de toutes sortes. L'essentiel, au final, est qu'elles soient en mesure de nous le rendre quand on le réclame. En l'occurrence, je comprends qu'il en va de même pour la CDC. D'ailleurs, j'appelle votre attention sur le taux de 5 % de reversement que nous proposons. On exige ainsi de la CDC un prudentiel de 95 %. C'est un record absolu et sans commune mesure avec les exigences de Bâle. Pour parler d'atteinte à la propriété, il faudrait que la Caisse fasse don du contrat d'un individu bien identifié. Mais, en l'espèce, nous sommes en présence d'un bien fongible. le reversement n'emporte aucun transfert de propriété des fonds sur un contrat déterminé, pas plus que l'argent de ses clients utilisé par une banque n'emporte dépossession de ceux-ci.

le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du samedi 14 novembre, le matin, l'après-midi et le soir, de la suite éventuelle du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Acte est donné de cette demande. Au vu du nombre d'amendements restant à examiner, nous pourrions également d'ores et déjà ouvrir la nuit du vendredi 13 novembre. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. Par ailleurs, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement sollicite du Sénat l'inscription de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 à l'ordre du jour du vendredi 20 novembre, le matin. à l'ordre du jour du vendredi 20 novembre, le matin. Nous pourrions fixer le début de l'examen de ce texte à onze heures et la durée de la discussion générale à quarante-cinq minutes. Y a-t-il des observations ?